Cet amendement a pour objet de compléter le code de la santé publique et le code pénal s'agissant des personnes atteintes d'une pathologie pour laquelle l'existence d'un risque accru de décès ou d'invalidité n'est pas scientifiquement démontrée, en particulier dans leurs conditions d'accès au crédit. Alors qu'il est prouvé depuis plusieurs années que, grâce aux traitements disponibles, l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH est identique à celle de la population générale, celles-ci continuent de se voir appliquer la surprime maximale de 100 % de leur assurance. Dès lors, on peut envisager que les organismes d'assurance soient tenus d'apporter la preuve de la justification médicale et scientifique des cotisations supplémentaires qu'ils entendent facturer aux personnes présentant un risque aggravé de santé. L'objet de cet amendement est donc de mettre fin à une pratique concernant certains emprunteurs potentiels qui n'apparaît plus justifiée au regard de l'état actuel de la médecine. La

; supprimer le plafond d'emprunt pour les personnes bénéficiant de la convention Aeras, c'est-à-dire en rémission depuis moins de cinq ans. À l'issue des travaux législatifs de l'Assemblée nationale, l'article 7 ne permet toujours pas aux signataires de cette convention de négocier sur la possibilité d'en appliquer les bénéfices à de nouvelles pathologies et sur la possibilité de réduire le délai du droit à l'oubli, au détriment des personnes concernées et de leurs projets. Pourtant, en matière de droit à l'oubli, le Gouvernement s'était engagé à ramener le délai à cinq ans après la fin du protocole de guérison, afin de permettre aux personnes ayant été atteintes d'une pathologie cancéreuse d'accéder à l'assurance emprunteur. Le Gouvernement a d'ailleurs rappelé cet engagement le 19 octobre dernier, à l'Assemblée nationale, sans néanmoins amender ce texte,

et insupportable que des personnes guéries ne puissent tourner la page de leur maladie et se lancer dans un projet de vie dans des conditions normales. Être constamment réduit à son ancienne maladie constitue une grande souffrance morale- et je

Ces amendements identiques témoignent d'une véritable convergence de vues sur la nécessité de faire enfin évoluer la loi sur ce sujet. Je m'en réjouis ! Je rappelle, par ailleurs, que les dispositions proposées s'appliqueront aux prêts qui ne sont pas déjà couverts par la suppression du questionnaire médical, cette suppression

parle d'expérience -c'est là l'assurance que les évolutions resteront tardives et lentes. Toutes les associations de patients que nous avons entendues dans le cadre de nos travaux concluent à l'incapacité de la convention Aeras à régler le problème de l'accès à l'assurance emprunteur dans des conditions normales pour les personnes malades ou guéries.

pour les plus fragiles, les malades, les célibataires et les plus âgés. Nous nous adressons à ceux qui, ayant obtenu un crédit,

Les associations que nous avons reçues considèrent que la santé ne peut être un objet de discrimination, ce en quoi elles ont parfaitement raison. Reste qu'il est aussi de notre devoir d'entendre l'ensemble des acteurs : certains s'opposent fermement à cette suppression, avec des arguments que nous pouvons recevoir. Aussi imparfaite soit-elle, la grille de référence Aeras apparaît comme un progrès pour l'accès des personnes les plus fragiles à l'emprunt. Les discussions doivent se poursuivre pour réduire les délais concernant le droit à l'oubli et étendre celui-ci à d'autres pathologies que les pathologies cancéreuses. En l'état des discussions, il est prématuré de supprimer le questionnaire de santé, même sous conditions.

et lever les obstacles auxquels doivent faire face les consommateurs pour changer d'assurance emprunteur. Une loi de 2017 a ainsi introduit la faculté de résiliation annuelle de l'assurance emprunteur, mais les consommateurs se sont rapidement heurtés à des difficultés qui ont eu pour conséquence de rendre ce droit peu effectif. Les rapporteurs Daniel Gremillet et Jean-Baptiste Blanc, dont je salue ici le travail, ont fait le choix de renforcer le droit existant. Ils ont réintroduit le dispositif qui avait fait l'objet d'un consensus entre députés et sénateurs, avec le soutien du Gouvernement,

de demander aux banques de motiver leur refus de résiliation, le cas échéant, et de renforcer la communication des banques auprès de leurs clients sur leur droit de résiliation, ainsi que sur la procédure qu'ils doivent suivre. La résiliation à tout moment que proposait ce texte issu de l'Assemblée nationale ferait courir un risque de démutualisation trop important. C'est un mouvement qui a d'ailleurs déjà commencé avec l'ouverture à la concurrence, mais qui est contenu pour le moment : les tarifs ont ainsi augmenté de 30 % pour les plus de 55 ans, plus de 55 ans, selon le CCSF. La possibilité de résilier à tout moment l'assurance emprunteur conduirait à une plus forte segmentation du marché au détriment des plus fragiles et de leur possibilité d'accéder à la propriété.

L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Madame la présidente, madame la vice-présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle étape de la navette parlementaire de la proposition de loi visant à réformer l'adoption.

si possible de l'enrichir encore, et de nous projeter vers son adoption définitive et sa mise en oeuvre, tant elle est attendue par de nombreuses familles, de nombreux professionnels et tant elle profitera à de nombreux enfants. Les enfants à qui le texte profitera sont, bien entendu, ceux qui, malgré les améliorations successives de notre système d'adoption, sont encore trop nombreux à ne pas bénéficier du projet de vie qui, pourtant, pourrait répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Ce n'est en effet pas faire insulte à notre politique d'adoption, faite de nombreux contrôles et de vérifications nécessaires, que de dire qu'elle suscite des espoirs parfois déçus. C'est un système avec ses forces, ses succès, mais qui ne remplit pas encore entièrement

de dispositions claires permettant de donner une famille à chaque enfant qui n'en aurait pas ou dont la famille ne serait plus en mesure de s'occuper de lui. Ce manque constitue une terrible rupture d'égalité, dont les conséquences peuvent être lourdes sur le développement personnel, affectif, psychologique de l'enfant. C'est la force de ce texte que de rendre possible l'adoption de davantage d'enfants pour lesquels celle-ci représente un horizon souhaitable. bien l'objet de l'article 4 : permettre à des enfants qui étaient privés jusqu'à présent d'une telle possibilité d'être adoptés de manière plénière après 15 ans par leurs beaux-parents, lorsqu'ils sont pupilles de l'État ou lorsqu'ils ont été judiciairement déclarés délaissés et sont donc dans des parcours de fragilité qui n'étaient pas suffisamment pris en compte.

chiffres en première lecture - et permet de plus en plus de mettre fin au bon moment aux relations toxiques qui existent parfois- nous le savons -entre un enfant et ses parents.

d'un mineur âgé de plus de 13 ans ou d'un majeur protégé hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. C'est une mesure juste, simple, claire, sécurisante.

Cela passe avant tout par des règles claires, du type de celles que l'on retrouvera demain, grâce à ce texte. Celles-ci concernent d'abord les agréments, avec des conditions de candidature, de formation et d'accompagnement des futurs adoptants plus étoffées. Elles concernent ensuite la prohibition de l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et soeurs, afin d'éviter le brouillage des lignes générationnelles. Elles concernent enfin le consentement des uns et des autres ; nous aurons, je le crois, l'occasion d'en débattre tout à l'heure.

mais à sa juste place -, comme à l'international, en matière d'intermédiation des adoptions. La France a développé un système, celui de l'aide sociale à l'enfance, dont l'existence même signale la préoccupation collective de garantir une intervention, un regard, une garantie publique

puissent bénéficier des mêmes conditions de sécurité. Aucune situation ne peut justifier que certains enfants bénéficient du statut de pupille de l'État quand d'autres en seraient privés, quelles qu'en soient les raisons. Le statut de pupille de l'État est le plus protecteur pour les enfants. L'autre part d'ombre sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer ici a trait aux adoptions internationales illégales. Je connais la préoccupation d'un certain nombre d'entre vous sur cette question. J'ai annoncé que le Gouvernement lancerait des travaux afin de faire oeuvre de transparence, de clarté et d'objectivité sur ces histoires, qui concernent un nombre important de nos concitoyens.

Je souhaite que la démarche retenue puisse être clarifiée dans les prochaines semaines et que les travaux débutent avant la fin de ce mandat. Tel sera le cas. Le dernier objectif tient à l'importance du combat collectif que nous devons mener pour faire progresser les droits des familles, de toutes les familles, pour reconnaître leur diversité et pour répondre à leurs attentes. En ouvrant enfin l'adoption aux couples non mariés, ce texte est cohérent avec l'évolution de la société. Il reconnaît les attentes de nouveaux modèles familiaux tout aussi légitimes, portant tout autant de promesses que les autres. Il était temps, même si cela gênera peut-être un certain nombre d'acteurs opposés à plus d'inclusion dans notre société. à la bioéthique, le texte apporte une solution adaptée aux difficultés rencontrées par certaines femmes ayant eu recours, avec l'entrée en vigueur de cette loi, à l'assistance médicale à la procréation (AMP) à l'étranger. Il le faut : c'est dans l'intérêt de l'enfant. Mesdames,

Enfin, en renforçant la diversité des conseils de famille et en réaffirmant un certain nombre de principes déontologiques, le texte garantit une meilleure prise en compte de la spécificité des multiples modèles familiaux qui font la richesse de notre société. C'est indispensable. Mesdames, messieurs les sénateurs, à de très nombreux titres, les mesures du texte permettent d'ancrer fermement et définitivement l'adoption dans la protection de l'enfance et dans une modernité soucieuse du bien-être de tous les membres de notre société, en particulier des plus jeunes et des plus fragiles. Toutes ces dispositions sont pensées pour le seul bénéfice d'enfants pour qui l'adoption est un horizon synonyme d'épanouissement et de familles, pour qui celle-ci représente un horizon lumineux. De nombreux enfants l'attendent encore. De nombreuses familles sont prêtes à le faire. À nous de leur en donner enfin la possibilité. La parole

Un autre renoncement peut, me semble-t-il, être salué. Dans un premier temps, l'Assemblée nationale avait totalement réécrit des pans entiers du code de l'action sociale et des familles, alors même que

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous revenons donc en cette fin de session parlementaire

lecture. En outre, il nous manque toujours l'avis du Conseil d'État et une étude d'impact sur ce projet de loi déguisé. Au vu des divergences entre nos assemblées, ces documents auraient pu utilement éclairer nos travaux. Pis, l'habilitation à légiférer par ordonnances, que nous avions supprimée en première lecture, a été rétablie par l'Assemblée nationale, ce qui nous semble particulièrement scandaleux alors que nous examinons une proposition de loi, et non un projet de loi. Le débat n'aura pas été sans heurts, comme en témoignent l'absence de compromis en commission mixte paritaire et les divergences qui demeurent entre nos deux assemblées sur des points essentiels. Nous sommes bien loin de l'esprit consensuel qui devrait nous animer afin de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel est toujours d'avoir une famille, comme le rappelle le rapport Limon-Imbert. Cette proposition de loi nous interroge également, car, loin de constituer une réforme globale de l'adoption, elle ressemble à un patchwork de mesures diverses aux enjeux aléatoires : diminution de l'âge des adoptants et de la durée de vie commune nécessaire, écart d'âge maximal entre l'adopté et l'adoptant, consentement pour l'adjonction du nom, sécurisation du statut des jeunes pupilles, etc. La mesure la plus emblématique de ce texte demeure l'ouverture du droit à l'adoption aux couples non mariés, qu'ils soient en concubinage ou liés par un PACS. Nous sommes favorables à une telle mesure, qui va dans le sens des évolutions sociétales et libère l'adoption du carcan d'une vision réductrice de la famille. Cette mesure répond ainsi ainsi à une exigence légitime d'égalité de droits et de liberté de choix. Pour autant, nous aurions souhaité que ce texte manie autant les symboles que les dispositifs opérationnels. Or il reste anecdotique face aux enjeux de l'adoption aujourd'hui. trop d'enfants se retrouvent encore sans famille. Fin 2019, 10 263 agréments étaient en cours de validité. Il y avait parallèlement 3 248 pupilles de l'État, et seuls 706 ont pu été adoptés, soit un peu plus de 20 %. Je rappelle que 49 % des enfants pupilles, pour lesquels le projet de vie est un projet d'adoption, n'ont pas été adoptés, le conseil de famille n'ayant pas réussi à leur trouver une famille, notamment au regard de leurs difficultés. Au regard de ces chiffres, Au regard de ces chiffres, ce n'est pas le changement de la composition du conseil de famille opéré par le texte qui résoudra le problème. On mesure ainsi les progrès à réaliser et le décalage entre ce texte et les véritables enjeux de modernisation de la procédure d'adoption, tant à l'intérieur Alors que les départements jouent un rôle décisif dans ces procédures, cette proposition de loi n'aborde qu'à la marge ce sujet. Nous estimons ainsi que la première urgence reste tout simplement d'appliquer le droit positif, notamment la loi du 14 mars 2016. Faute de moyens, on constate une grande iniquité territoriale. Nous jugeons finalement maladroite la volonté de revenir, au détour de cette proposition de loi, sur les débats concernant la bioéthique. Ce sujet mérite mieux que des débats à la hussarde. Malheureusement, ce point relatif à l'adoption des enfants nés d'une PMA a constitué le principal point de blocage entre nos assemblées, loin de l'esprit du rapport Limon-Imbert. Enfin, ce texte soulève de grandes incompréhensions et de grandes résistances, notamment chez les professionnels du droit ; ces obstacles ne sont pas totalement levés aujourd'hui. Le groupe communiste

mes chers collègues, ce texte part d'un constat que nous partageons tous : le régime juridique de l'adoption a des lacunes qu'il faut combler. En ce sens, le rapport de nos collègues

de trop nombreuses familles veulent adopter sans trouver de solutions, et de trop nombreux enfants restent sans famille. En outre, le principal sujet a changé. Quand on parle d'adoption, c'est non plus la famille adoptante qui prime, mais bien l'enfant. C'est sur lui que doit se concentrer notre attention, c'est lui que nous devons placer au coeur de nos dispositifs. Nous devons offrir à cet enfant une famille qui l'aidera à grandir et à se développer harmonieusement.

Les objectifs sont simples : mieux préparer les familles à l'adoption, notamment au regard des profils des enfants adoptables, faciliter l'adoption des enfants qui peuvent l'être, au besoin sous une forme simple, mieux former les parties prenantes de l'adoption. Ce texte, que l'on pourra juger inabouti, comporte néanmoins de bonnes mesures. Tout d'abord, l'élargissement de l'adoption au concubinage et au PACS permet d'ouvrir l'adoption à un public plus large. Dans le même temps, afin de fluidifier les procédures, le tribunal pourra prononcer l'adoption de mineurs de plus de 13 ans ou de majeurs protégés lorsqu'ils sont hors d'état d'y consentir.

Je sais que cette disposition a fait débat, mais je reste convaincue que cet accompagnement est nécessaire, tant pour protéger les adoptants contre divers risques que pour lutter contre des dérives que l'on a pu connaître dans certains pays, avec une véritable exploitation du corps de la femme. Il n'est qu'à se rappeler l'histoire des fermes à bébés, mes chers collègues ... Ce texte apporte également des dérogations à l'interdiction de l'adoption plénière des mineurs de plus de 15 ans ans pour les enfants du conjoint, les pupilles de l'État ou des enfants déclarés judiciairement délaissés. C'est, je le crois, une mesure pleine de bon sens, qui permet de s'adapter à la réalité des familles d'aujourd'hui. Cette proposition de loi entend aussi faciliter l'adoption simple, majoritaire en France, qui concerne bien souvent un majeur et qui est majoritairement réalisée dans un contexte intrafamilial. Le Sénat a supprimé la période de placement obligatoire pour les majeurs dans ce cas. En effet, il s'agit souvent d'adultes qui connaissent leur adoptant et qui ont souvent déjà un toit.

S'il est urgent de faciliter les adoptions, il faut aussi que le désir d'avoir un enfant se plie au principe de l'intérêt supérieur de ce dernier. Malgré les désaccords qui ont pu perdurer au cours de la navette parlementaire, la protection de l'enfant a été au coeur de nos débats. Plusieurs mesures vont dans le bon sens.

La préparation à la parentalité des futurs adoptants va également dans le sens de l'intérêt de l'enfant. La généralisation, dans tous les départements, de l'obligation de formation au profit des membres du conseil de famille était très attendue. De manière générale, toute aide à la parentalité, moment compliqué pour tous les parents, adoptants ou non, ne peut être que bénéfique. Enfin, nous apportons tout notre soutien à l'amélioration du statut des pupilles de l'État. En ce qui concerne

Je tiens à saluer l'esprit constructif de la commission des lois, qui a consenti de nombreuses concessions, comme Mme le rapporteur l'a rappelé. Nous nous opposons néanmoins à la suppression de l'article 9 visant à établir la filiation de la mère d'intention dans le cas d'une AMP réalisée à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi relative Nous soutiendrons donc l'amendement du Gouvernement. Il est incontestablement dans l'intérêt de l'enfant que la deuxième personne puisse l'adopter, y compris si la mère biologique Même si elle n'a pas porté l'enfant, elle dispose le plus souvent d'un vécu commun avec ce dernier, dans le cadre d'un projet familial conçu à deux. Des conflits entre adultes n'ont à avoir de répercussions ni sur la filiation, qui constitue un acte social, ni sur les liens affectifs. Cette disposition reste encadrée, puisque son application requiert une opposition de la mère biologique « sans motif légitime ». Il reviendra au juge de statuer au cas par cas, dans l'intérêt de l'enfant. Faisons-lui confiance

: « Dans les faits, et bien que les outils existent, le devenir à long terme de l'enfant protégé est donc rarement pris en compte en France, où la priorité est celle du maintien des liens avec les parents à tout prix.

Le parcours du combattant des adoptants ne sera pas plus allégé, laissant les enfants dans une longue période d'incertitude. Pour que l'enfant puisse être adopté, encore faut-il qu'il soit adoptable. ne faut pas précipiter les choses en toutes circonstances, mais il n'est pas inutile de les simplifier lorsque les conditions sont réunies. Surtout, il convient de consacrer à cette politique les moyens qu'elle mérite.

Je la salue et lui souhaite un prompt rétablissement. Chaque année, 950 enfants sont adoptés dans notre pays. C'est peu, alors que l'on compte 2 700 pupilles de l'État et 14 000 agréments accordés à des familles pour accueillir et élever un enfant. Par conséquent, cette proposition de loi tente d'apporter des réponses à cette situation humainement difficile. Sur ce point, le texte contient plusieurs avancées que le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain tient à saluer. Au stade de la première lecture, nous avions regretté l'absence de vision globale sur la protection de l'enfance,

il aurait été bienvenu de faire le bilan de la mise en oeuvre du droit existant, en particulier de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance, comme des dispositions de la loi de 2002 relative à l'accès aux origines des personnes bénéficiaires accèdent cette année à la majorité. En revanche, nous avions salué dans ce texte une mesure phare que nous avons portée et défendue, à savoir l'élargissement de l'adoption aux personnes liées par un PACS ou en concubinage, qui a été approuvé par la commission des lois après un débat nourri. L'ouverture du droit à l'adoption pour les couples pacsés ou en concubinage accompagne les évolutions de notre société, prenant acte, en quelque sorte, qu'il existe non pas un seul modèle familial, mais des familles plurielles, qui ont pour dessein la stabilité et la protection des enfants. Ainsi, l'exclusion de certaines familles de la possibilité d'adopter en raison de leur composition ou de leur statut conjugal n'existera plus sur le plan légal. C'est tant mieux. toutefois, avec les familles homoparentales, le chemin qui reste à parcourir dans certaines mentalités, dans certains cénacles, chez certains membres des conseils de famille pour accompagner accompagner cette avancée. Là encore, la promulgation de la loi ne saurait à elle seule réaliser ce progrès. L'État devra s'assurer de son application et de l'absence de comportements discriminatoires. Un autre point du texte nous paraît important : l'idée de valoriser l'adoption simple pour permettre aux enfants adoptés de conserver le lien d'origine de leur filiation ainsi que leurs droits au sein de leur famille biologique. il nous paraît important de veiller à ce que le consentement des familles qui confient leur enfant soit éclairé. Sur cet aspect, la rédaction proposée renforce les parents biologiques : ces derniers ont désormais la possibilité d'être accompagnés de la personne de leur choix afin de consentir à l'adoption, le consentement étant toujours recueilli par procès-verbal. Je considère qu'il s'agit d'un acte protecteur pour l'enfant ainsi remis à l'aide sociale à l'enfance afin d'être admis en qualité de pupille.

dans le cadre d'une séparation. Au-delà de ces points d'accord, un point de désaccord majeur demeure avec la majorité de l'Assemblée nationale : celui du rétrécissement de l'activité des OAA. Nous défendons la possibilité pour les familles de conserver une alternative à l'aide sociale à l'enfance pour confier leur enfant à l'adoption, en maintenant la possibilité pour les OAA de recueillir un enfant en France en vue de l'adoption.

question., indépendamment des quelques amendements que nous proposons, qui relèvent plus de la clarification que de questions de fond, nous souscrivons au plus grand nombre des dispositions de ce texte. sont parfois techniques, mais leur portée humaine est forte et elles répondent aux attentes de notre société, des enfants et des familles. Pour ces raisons, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera en faveur de cette proposition de loi.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j'associe à cette intervention mon collègue Xavier Iacovelli. Nous voici de nouveau réunis pour examiner, en nouvelle lecture, la proposition de loi de notre collègue députée Monique Limon visant à réformer l'adoption. l'adoption. Fruit d'un travail transpartisan, ce texte répond à des objectifs que nous partageons pleinement : sécuriser le recours à l'adoption, avec le souci de donner une famille à l'enfant, et non l'inverse, renforcer également également le statut de pupille de l'État, en partant de l'intérêt supérieur de l'enfant. En première lecture, le texte a fait l'objet de modifications importantes de la part de notre rapporteur, dix articles ayant été supprimés. Nos débats ont toutefois permis de conserver certaines avancées importantes du texte, notamment l'ouverture de l'adoption plénière aux concubins et aux couples pacsés, pacsés, le principe d'un écart d'âge maximum de 50 ans entre l'adoptant et l'adopté, le renforcement de la formation et de la préparation des membres des conseils de famille et des candidats à l'adoption, l'amélioration de la prise en compte de la situation de l'enfant. Nous avons également pu rétablir en séance, dans un objectif de sécurisation, l'interdiction des adoptions internationales individuelles. Si la commission mixte paritaire a échoué, les travaux de nos deux assemblées en nouvelle lecture ont permis des compromis que je souhaite saluer. La commission des lois a conservé un nombre important de dispositions réintroduites par l'Assemblée nationale. Celles-ci permettent de répondre aux objectifs du texte et sont pour certaines le fruit de rédactions de compromis que notre groupe a défendues en première lecture. Je pense à l'extension des possibilités d'adoption plénière des enfants âgés de plus de 15 ans, essentielle pour favoriser l'adoption des pupilles de l'État et des enfants déclarés délaissés. Je pense Je pense également au meilleur encadrement de la délivrance des autorisations aux OAA pour l'adoption internationale, cohérent avec les objectifs de sécurisation et de prévention des pratiques illicites. Nous nous en félicitons. Je pense, enfin, à l'interdiction explicite de l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et soeurs, tout en ménageant une dérogation conforme à l'intérêt de l'adopté. Je veux ici saluer l'esprit de consensus qui a guidé les travaux de notre rapporteur dans cette nouvelle lecture. Au-delà des clivages qui traversent cet hémicycle, objectif commun est de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant et de sécuriser le recours à l'adoption. Certes, des points de désaccord persistent. le cas de la suppression du dispositif transitoire d'établissement de la filiation des enfants nés par recours à l'AMP à l'étranger par un couple de femmes, alors même que celui-ci permet de garantir l'intérêt de l'enfant en permettant de sécuriser sa filiation. sa filiation. De même, la faculté pour les OAA de recueillir des enfants pour l'adoption nationale comporte à notre sens un risque de dérives et s'inscrit en décalage avec l'objectif de renforcement du statut protecteur de pupille.

Au 31 décembre 2019, plus de 10 000 agréments étaient en cours de validité, mais 706 pupilles de l'État seulement sur les 3 248 recensés ont été adoptés. Trop d'enfants sont encore laissés sur le bord du chemin menant à l'adoption. Ce constat nous montre l'urgente nécessité de combler les lacunes juridiques de notre droit positif. La proposition de loi que nous examinons ce soir en nouvelle lecture a pour objectif de refonder le modèle de l'adoption afin de permettre à chaque enfant de trouver le projet de vie le plus adapté et le plus sécurisant pour lui. À cet égard, je souhaite exprimer deux regrets au nom du groupe Les Indépendants- République et Territoires. En premier lieu, nous touchons, avec ce texte, à un sujet majeur et extrêmement sensible. Une initiative du Gouvernement par le dépôt d'un projet de loi aurait été préférable à une proposition de loi qui nous prive d'une étude d'impact et de l'avis du Conseil d'État. En second lieu, nous ne sommes pas parvenus à un texte de compromis lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Celle-ci a achoppé sur une seule disposition : l'article 9 . Au cours de l'examen du texte en commission en nouvelle lecture, le Sénat est revenu avec pertinence sur certaines mesures problématiques adoptées par nos collègues députés. Je pense tout d'abord aux conditions d'âge et de vie commune s'imposant aux couples candidats à l'adoption, figurant à l'article 2. Sur ce point, le Sénat s'était unanimement positionné, en première lecture, en faveur du maintien du droit en vigueur. Or l'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, l'assouplissement de la durée de la communauté de vie,

de recueillir des enfants en France en vue de l'adoption, souhaitant conférer ainsi un monopole à l'aide sociale à l'enfance. Nous ne partageons pas cette position. Bien au contraire, ces organismes constituent une alternative intéressante à l'ASE. Leur activité est encadrée et bénéfique pour tous. Là encore, nous préférons nous en tenir au droit en vigueur.

sans motif légitime » de faire une reconnaissance conjointe rétroactive pour établir la filiation de la mère d'intention. Il donne la possibilité à celle-ci de demander à adopter l'enfant dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi. l'appréciation du « motif légitime », trop floue, est source d'insécurité juridique. Cet article semble finalement n'avoir pour objectif que de régler un litige entre adultes, sans prendre en considération l'intérêt de l'enfant. Avant de conclure, je tiens à saluer la qualité des travaux et l'implication tout au long des débats de Mme le rapporteur, Muriel Jourda.

Ce texte, qualifié de décevant par les acteurs de la protection de l'enfance, apparaît à certains égards dogmatique, alors même que le sujet, tout le monde en convient, est très sensible, voire parfois douloureux, pour bon nombre d'enfants Toutefois, la commission s'est efforcée de l'examiner, à chacune de ses lectures, sans jamais perdre de vue l'intérêt supérieur de l'enfant, et avec la ferme volonté de s'en tenir à une vision purement réaliste, en s'appuyant notamment sur les retours des associations et des acteurs de la protection de l'enfance. C'est dans cet état d'esprit que nous avons souhaité maintenir le droit en vigueur à propos des critères requis pour qu'un couple puisse entamer la procédure d'adoption. En effet, il nous est apparu que l'assouplissement de ces critères voulu par l'Assemblée nationale s'affranchissait complètement de la réalité des situations des familles qui souhaitaient adopter. Avec ce même pragmatisme, la commission vous propose également de maintenir la possibilité pour les organismes agréés d'accueillir des enfants en vue d'une adoption. Sur ce sujet si délicat, qui concerne le devenir de plusieurs milliers d'enfants, il est en effet souhaitable, et même essentiel, de maintenir une autre solution que l'aide sociale à l'enfance, tout en reconnaissant que ces organismes ne peuvent être exemptés d'un contrôle strict

de demander la possibilité de légiférer par ordonnances sur un sujet aussi sensible. Le texte actuel n'est-il pas une vraie occasion de débat et de réforme ? Si le Gouvernement souhaite aborder d'autres modifications s'agissant de l'adoption, pourquoi ne pas les présenter, de la manière la plus transparente possible, dans le cadre de l'examen de ce texte ? J'ai été choqué, mais pas étonné, puisque cette méthode est révélatrice de l'état d'esprit d'un Gouvernement qui fait vraiment tout son possible pour s'affranchir s'affranchir des débats parlementaires, pourtant au coeur de l'équilibre de nos institutions. À cet égard, je ne peux que m'associer à la position de notre rapporteur, Muriel Jourda, et de notre collègue Laurence Harribey.

l'adoption de l'enfant par la mère d'intention, y compris quand la mère biologique « s'y oppose sans motif légitime ». Au-delà du caractère assez flou de la notion de motif légitime, cela ne revient-il pas tout simplement à priver la mère biologique de son droit au consentement à l'adoption ? Cette disposition ne concerne d'ailleurs pas directement l'enfant, puisqu'il s'agit d'un litige entre deux personnes adultes. C'est à ces deux titres que la commission des lois a réitéré sa ferme intention de supprimer cette disposition qu'elle juge inadaptée, dans la mesure où elle n'a pas pour objectif premier l'intérêt supérieur de l'enfant. mes chers collègues, j'y insiste, notre groupe restera ferme sur les apports de la commission des lois, dont certains font l'objet d'un large consensus, nourri par l'attachement général à défendre l'intérêt supérieur de l'enfant.

l'équilibre affectif et psychologique d'un enfant étant évidemment sans lien avec statut marital de ses parents. D'autres articles ouvrent l'adoption plénière à des enfants de plus de 15 ans, qui étaient privés jusqu'à présent de cette possibilité.

été adoptés, plus de trois enfants sur quatre se retrouvant sans solution. Ce texte est néanmoins insuffisant à plusieurs égards : pas d'amélioration de la situation des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance ; pas d'avancée sur l'accès aux origines des enfants nés dans le secret et admis de ce fait au statut de pupille de l'État

Ce dispositif est évidemment protecteur pour l'enfant, et ce pour une raison très simple : un enfant ne devrait pas se voir privé d'un parent simplement à cause des conditions dans lesquelles ses parents se sont séparés.

Imaginez une seconde ce refus appliqué aux couples hétérosexuels : franchement, qui, ici, pourrait s'opposer à ce qu'un père puisse être reconnu comme tel simplement parce que la mère, dont il s'est séparé avant la naissance, n'y consent pas ? Vous nous dites que nous sommes dogmatiques,

Surtout, cette disposition est quand même très encadrée, l'article 9 disposant que « le juge prononce l'adoption s'il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige

nous qui serions dogmatiques ? Honnêtement, je ne vous suis pas. En ce qui nous concerne, au groupe Écologiste -Solidarité et Territoires, pas d'ambiguïté, nous voterons l'amendement du Gouvernement demandant le rétablissement de l'article 9 .

quand le Président de la République a nommé un secrétaire d'État à la protection de l'enfance : comment se fait-il que, sur une politique qui relève à 100 %

en commission, j'ai envie de saluer votre engagement. Ce que vous avez fait dans votre ministère a montré toute votre volonté sur ce sujet difficile.

L'idée est simplement de corréler au maximum les conditions « naturelles » et « adoptives ». Sans parler d'adoption, on peut devenir parents après un an de communauté de vie,

L'avis de la commission est défavorable. Effectivement, la notion de discernement est utilisée en droit de la famille, mais jamais comme critère justifiant qu'un enfant puisse donner son consentement. Un enfant donne son avis lorsqu'il est capable de discernement, ce qui reste à l'appréciation du juge. rien n'interdit au juge d'entendre l'enfant de 13 ans pour avoir son avis, mais le discernement n'est pas un critère de consentement ; c'est un critère d'avis. Le consentement est fixé à un âge, certes arbitraire, mais cela paraît plus raisonnable dans l'architecture du droit de la famille. Quel est l'avis

C'est un dispositif transitoire, très encadré, comme l'ont rappelé certains d'entre vous, pour régler la situation de ces couples de femmes qui ont eu recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger et qui se sont séparés depuis le projet parental commun. Mais il y avait bien un projet parental, et c'est ce qui compte. Il s'agit d'un mécanisme exceptionnel, j'y insiste. La simple opposition de la femme qui a accouché ne peut suffire, et le juge doit s'assurer que son refus n'a pas de motif légitime. Si tel est le cas, le juge établit le lien de filiation à l'égard de la seconde femme. En d'autres termes, l'adoption ne sera prononcée que si ce refus n'est pas légitime et si, bien évidemment,

la filiation est établie si elle correspond à une réalité. Si tel n'est pas le cas, elle peut être contestée. C'est là, me semble-t-il, que la discrimination pourrait intervenir, c'est-à-dire entre deux parents, hétérosexuels ou homosexuels, dont l'un ne serait pas le vrai parent biologique : à l'un on refuserait un lien adoptif, tandis qu'on l'autoriserait à l'autre. Or, dans un couple hétérosexuel, un homme qui voudrait se déclarer le père alors qu'il ne l'est pas devrait adopter. En aucune façon, on ne forcerait la mère

secrétaire d'État. Je me permets de préciser que le Gouvernement n'a pas cherché à rétablir tout ce qui avait été supprimé par le Sénat ... Le Sénat non plus

s'agit de réintroduire l'interdiction du recueil direct d'enfants en France par les organismes autorisés pour l'adoption, les fameux OAA. Cette interdiction, je vous le redis, est conforme à l'intérêt de l'enfant, car elle garantit que tous les enfants privés définitivement de la protection de leur famille d'origine bénéficieront du statut de pupille de l'État. Or c'est le statut le plus protecteur pour les enfants.

sur l'accompagnement, des départements notamment, en matière d'adoption des enfants à besoins spécifiques. D'ailleurs, dans votre texte, vous consacrez cette expertise.

qui prévoit expressément dans son article 11 que les départements peuvent prendre appui sur ces associations dans la recherche de familles adoptantes pour des pupilles pour lesquels un projet d'adoption est souhaité. Nous souhaitons donc conforter les OAA en France sur cette mission-là, mais nous souhaitons aussi

des mineurs en vue de l'adoption par les organismes autorisés pour l'adoption en France. La majorité des acteurs de la petite enfance s'accorde à reconnaître l'importance d'un accompagnement après l'adoption à la et de ses parents adoptifs pour la réussite du projet parental, mais le caractère obligatoire prévu dans la proposition de loi initiale est contesté. En effet, dès lors que l'adoption est prononcée, y compris en vertu d'une décision étrangère, les adoptants sont des parents de plein exercice et l'intervention d'un tiers ne devrait pas pouvoir leur être imposée autrement que sur décision d'un juge, en cas de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant. Cet accompagnement post-adoption, qui ne serait obligatoire qu'en cas d'adoption internationale,

d'une décision étrangère. Pourtant, cet accompagnement nous semble essentiel, car il permet d'apporter une aide, des conseils, dans les premiers temps de découverte et d'affiliation entre l'enfant placé en vue de l'adoption ou adopté et ses parents. Par ailleurs, le pupille placé en vue de l'adoption reste sous la responsabilité du tuteur et du conseil de famille jusqu'au prononcé de l'adoption. Il revient à ces derniers de s'assurer de la bonne intégration de l'enfant au sein de sa famille adoptive et, le cas échéant, de prendre toutes les mesures qui seraient nécessaires si des difficultés venaient à apparaître.

des pays d'origine, chaque adoptant prenant un engagement moral auprès de ces derniers, qu'il nous revient de garantir à leurs côtés dans le cadre des relations que nous entretenons avec ces pays.

est parfois nécessaire, notamment pour les professionnels, de clarifier les choses afin que le droit soit bien appliqué. À l'heure actuelle en effet, le code de l'action sociale et des familles prévoit que les parents sont invités à consentir à l'adoption lorsqu'ils remettent leur enfant à l'aide sociale à l'enfance en vue de son admission au statut de pupille de l'État, mais l'article

Inversement, ce n'est pas parce que les parents ont consenti à l'adoption de leur enfant lorsqu'ils l'ont remis à l'aide sociale à l'enfance que ce dernier sera nécessairement adopté. Pour cela, il est nécessaire que le conseil de famille prenne une décision en ce sens. En conclusion, la rédaction actuelle du code de l'action sociale et des familles produit les mêmes effets juridiques que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, mais induit les parents en erreur sur la réalité de leurs droits et contribue ainsi à alimenter l'idée que le statut de pupille de l'État a pour seul objectif de déboucher sur une adoption. Or l'adoption peut ne pas être dans l'intérêt d'un pupille de l'État, par exemple lorsque l'enfant a tissé des liens forts avec sa famille d'accueil ou lorsqu'il ne souhaite pas être adopté.

le contraire ! Les parlementaires ont ainsi ajouté un certain nombre de dispositions qui permettent d'éclairer le consentement des parents au moment où celui-ci est exprimé et de ne pas les entretenir dans l'illusion que le consentement qu'ils donneraient en première intention pourrait être renversé par une absence de consentement au moment de l'adoption. Pour toutes ces raisons, il nous semble important que cet article 13 puisse être rétabli dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

En ce qui concerne la gouvernance de la vie de l'enfant, il a laissé le législatif au conseil et l'exécutif au tuteur, celui-ci étant le représentant légal de l'enfant. Il apparaît donc discutable que, demain, l'ensemble des pouvoirs puissent être concentrés entre les mains du tuteur, lui offrant en outre la possibilité d'être élu président du conseil de famille et d'avoir voix prépondérante en cas de partage des voix, ce qui n'aurait pu être le cas dans la tutelle de droit commun, où le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Pour respecter, dans l'intérêt des enfants pupilles, la philosophie même de la tutelle, le partage nécessaire des prérogatives de l'un et de l'autre, le présent amendement tend à s'aligner sur la tutelle de droit commun, ce qui correspond au dispositif du code civil.

Mme Michelle Meunier. Dans la tutelle de droit commun, le tuteur ne vote pas. En effet, depuis 2007, le législateur a entendu préserver les rôles distincts des deux organes de la tutelle. En ce qui concerne la gouvernance de la vie de l'enfant, il a laissé le législatif au conseil et l'exécutif au tuteur, celui-ci étant le représentant légal de l'enfant. Il ne nous apparaît donc pas judicieux, si le présent texte devait être adopté en l'état, que l'ensemble des pouvoirs puissent être concentrés entre les mains du tuteur, lui offrant en outre la possibilité d'être élu président du conseil de famille et d'avoir voix prépondérante prépondérante en cas de partage des voix, ce qui n'aurait pu être le cas dans la tutelle de droit commun, où le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose donc de conserver le droit en vigueur : le tuteur est présent au

sociale. Il est à mon avis difficilement compréhensible que la défense des postulants à l'adoption se fasse à l'intérieur des conseils de famille, au détriment des enfants, privant ces derniers du regard et de l'expertise d'un psychiatre, d'un conseiller d'éducation, d'un juriste ou même d'un ancien responsable d'une maison d'enfants. Ces deux personnes qualifiées vont participer à la définition du projet de vie de l'enfant pupille de l'État, en prenant en compte leurs besoins spécifiques. Cet amendement a également été travaillé avec Enfance et familles d'adoption.

compétente en matière de protection de l'enfance et en matière médicale, psychologique ou sociale et une personne compétente en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations. Un tel équilibre nous semble nécessaire. Nous